Or la tension sur les prix agricoles pourrait avoir pour effet, si l'on encourageait les méthanisations, l'abandon d'une agriculture nourricière, d'une agriculture de fourrage, dont l'objet est de nourrir les êtres humains et les animaux.

pour objet d'éviter que des projets à caractère industriel ne s'implantent dans des zones agricoles en portant de 50 % à 80 % le taux d'intrants permettant de considérer un projet de méthaniseur comme nécessaire à l'activité agricole. Je suggère donc le retrait de

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable

Cet amendement vise à rétablir l'interdiction pour une installation de production de biogaz de cumuler le dispositif de certificat de production de biogaz avec un dispositif de soutien à la production d'électricité à partir de biogaz. Dès lors qu'une nouvelle source de revenus est introduite, comme cela serait le cas avec les certificats de production de biogaz, il serait nécessaire de modifier les autres dispositifs de soutien pour les prendre en compte et de procéder à une nouvelle notification auprès de la Commission européenne au titre de l'encadrement européen des aides d'État.

effets, ou loi Climat et résilience, de ce dispositif de soutien extrabudgétaire, destiné à compenser les baisses des tarifs d'achat. Le texte issu des travaux de la commission corrige une iniquité sans induire de surrémunération. En effet, il est curieux de ne pas appliquer un même dispositif de soutien extrabudgétaire au biogaz selon qu'il est utilisé en cogénération ou en injection. C'est contraire au principe de neutralité technologique. De plus, l'article L. 446-92 du code de l'énergie prévoit que les modalités d'application des certificats de production, notamment les catégories et les volumes, sont déterminées par arrêté du ministre de l'énergie, après avis de la Commission de régulation

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de réaliser de manière anticipée des investissements de renforcement des réseaux de gaz naturel pour le raccordement d'installations de production de biogaz. de biogaz. Il tend à préserver le cadre législatif en vigueur pour le dispositif d'aide au renforcement des réseaux de gaz naturel pour le raccordement d'installations de production de biogaz. Un tel dispositif nécessite en effet de trouver un équilibre entre le raccordement de nouvelles installations de production de biogaz et les coûts supportés par les utilisateurs des réseaux de gaz naturel. Il est donc important de préserver une validation des projets de renforcement par la Commission de régulation de l'énergie en amont de leur réalisation. La modification de l'article L. 453-9 du code de l'énergie pourrait rompre l'équilibre du dispositif d'aide au renforcement des réseaux, le risque étant de lancer de façon anticipée des projets de renforcement qui se révéleront peu

d'anticipation de la réalisation de travaux de raccordement par les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz. L'amendement n° 595 du Gouvernement vise à revenir sur cette simplification, pourtant très demandée par les porteurs de projets. L'amendement n° 575 rectifié tend au contraire à préciser que cette anticipation doit s'articuler avec les pouvoirs de la Commission de régulation de l'énergie, prévus notamment à l'article L. 453-2 du code de l'énergie. Il s'agit d'une demande légitime de cette autorité, dont l'expertise est incontestée en matière de régulation du marché du gaz.

En effet, l'enfouissement des déchets n'est pas une source renouvelable d'énergie. Nous avons voté dans la loi Agec la réduction de moitié des déchets enfouis d'ici à 2025. Dans cette perspective, la place des déchets organiques n'est plus du tout dans une décharge, mais dans un compost

qui resteraient considérés comme des énergies renouvelables. D'autre part, cela serait contraire à l'article 19 du projet de loi, qui a institué un cadre législatif précis pour le gaz bas-carbone, en lui appliquant par ailleurs un seuil strict d'émissions de gaz à effet de serre (GES). La commission demande le retrait de cet amendement.

ou, tout du moins, sans les myriades d'impuretés toxiques du gaz de décharge. Les collectivités doivent organiser la collecte des biodéchets d'ici à 2024. L'enfouissement et l'incinération des biodéchets vont baisser, et c'est heureux. raison de plus pour en finir avec l'aberration que constituent leur enfouissement et leur incinération. Brûler des déchets humides consomme presque autant d'énergie qu'en produire ; cela n'a aucun sens. La gestion de nos déchets représente 4 % de nos émissions de gaz à effet de serre ; c'est le quatrième poste d'émission après les transports, l'industrie et l'agriculture. Quel

Mes chers collègues, les mécanismes de garanties d'origine et de certificat de production, qui permettent au consommateur final de connaître la part de biogaz utilisée dans sa consommation, ne concernent, jusqu'à maintenant, que le seul biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel.

Cet amendement a donc pour objet d'étendre les garanties d'origine et les certificats de production au biogaz non injecté dans le réseau de gaz naturel, ce qui permettrait de mobiliser le gisement des exploitations agricoles trop petites ou trop éloignées des réseaux.

446-7 à L. 446-11 du code de l'énergie ; ne lui sont pas ouverts les dispositifs de soutien extrabudgétaires, comme les garanties d'origine et les certificats de production, ni les dispositifs expérimentaux, comme les contrats d'expérimentation. C'est la raison pour laquelle les trois amendements identiques visent à ouvrir les deux mesures de soutien extrabudgétaires à un tel usage du biogaz. Si je partage l'objectif des auteurs des amendements, la filière du biogaz non injecté me semble insuffisamment mature à ce stade pour envisager une évolution du cadre de régulation. De plus, l'esprit des amendements est pour partie satisfait, puisque les contrats de long terme sur le biogaz, que la commission a institués à l'article 18, dans un nouvel article L. 443-4-1 du code de l'énergie concernent bien la filière du biogaz non injecté. En effet, leur champ couvre l'approvisionnement en biogaz, gaz renouvelable ou gaz bas-carbone, quel que soit son usage. Enfin, aucune des personnes interrogées au cours de nos auditions, y compris les professionnels du biogaz,

En effet, on observe aujourd'hui que la mise en place d'installations agrivoltaïques dans nos territoires est réalisée au travers d'un contrat, entre les développeurs énergéticiens et les propriétaires terriens, un bail emphytéotique normalement prévu pour établir des contrats entre les agriculteurs et les propriétaires fonciers. Dans un deuxième temps, l'énergéticien propose à l'agriculteur un prêt à l'usage, mécanisme de droit privé sortant l'agriculteur du cadre très protecteur du fermage ou de l'emphytéose, prévus dans notre droit rural. Cette inversion historique est problématique à plusieurs égards. Même si le prêt à l'usage gratuit peut sembler avantageux, c'est un mirage, car les droits réels sur la parcelle sont détenus par les l'énergéticien bénéficiant du bail emphytéotique. Ce dernier peut, par exemple, avec un préavis de six mois, expulser l'agriculteur de la parcelle. Par ailleurs, le fait que l'agriculteur n'ait plus de lien direct avec le propriétaire foncier constitue une rupture dans la tradition agricole française et, pour nos petites exploitations agricoles familiales, L'introduction dans le code rural d'une nouvelle catégorie, le bail emphytéotique agrivoltaïque, s'imposant aux installations du même nom, fournit par la séparation des volumes du haut et du bas les garanties nécessaires, d'une part, à l'exploitant photovoltaïque et, d'autre part, à l'exploitant agricole. Il représente une sécurité

L'hydrogène renouvelable est un vecteur énergétique clé pour décarboner l'industrie et la mobilité, de surcroît dans le contexte d'urgence climatique et énergétique actuel. Le présent amendement vise à instaurer une mesure concrète permettant d'accélérer dès aujourd'hui la construction d'installations de production d'hydrogène renouvelable dans nos territoires. Il s'agit de permettre aux installations de production d'hydrogène renouvelable de participer à des opérations d'autoconsommation, notamment par le raccordement indirect des unités de production d'hydrogène renouvelable aux installations d'énergies renouvelables. Le déploiement de l'hydrogène renouvelable est essentiel pour la réindustrialisation, pour la souveraineté énergétique de la France et pour l'amélioration significative de la compétitivité économique des projets lancés par nombre de collectivités territoriales pour décarboner les transports publics et les sites industriels de leur territoire.

et L. 315-2 du code de l'énergie n'excluent pas par principe la possibilité pour un propriétaire de participer à de telles opérations. À l'inverse, le raccordement indirect, mentionné dans l'objet de l'amendement, est prohibé. De plus, les besoins de mutualisation pourront être couverts,

La suppression de l'article 17 aurait de nombreux effets de bord. D'une part, elle conduirait à abroger non seulement les contrats d'achat de long terme, mentionnés dans l'objet de l'amendement,

d'une ressource financière intéressante, car les contrats d'achat de long terme sont très demandés en cette période de crise. Notre commission- je tiens à le dire -a tenu à bien encadrer le dispositif des contrats d'achat de long terme. Nous avons exigé une autorisation de fourniture, en précisant son utilisation par les collectivités territoriales. veillé à ce que le soutien privé aux projets d'énergies renouvelables n'évince pas celui public, inscrivant directement l'accord préalable du porteur de projets et l'absence d'effet rétroactif sur les contrats

pour l'ensemble des consommateurs, quelles que soient leurs caractéristiques. Le problème majeur, c'est l'organisation du marché européen. C'est une affaire européenne. Nous attendons du Gouvernement et du Président de la République

». Pour quel résultat ? Une fragmentation du réseau des acteurs, qui empêchera la solidarité tarifaire

Le service public sera rendu pour ceux qui n'auront pas eu le choix de faire autrement, jusqu'à la prochaine crise. La Commission

Le scrutin est ouvert.

... Le scrutin est clos.

qui devra être fixée en fonction de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution. Enfin, il vise à remplacer la référence au « code des marchés publics », qui n'existe plus, par une référence au « code de la commande publique »

à M. Daniel Gremillet. Cet amendement a pour objet de consolider la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à des contrats d'achat de long terme d'électricité ou de biogaz.

n° 237 rectifié. Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats de vente directe à long terme d'électricité. En l'état, les règles de la commande publique, en particulier celles qui encadrent la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces contrats. ces contrats. Il s'agit ici en particulier de faire corréler la durée du contrat avec celle de l'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, et ce y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquièrent pas ces installations. En effet, la nature spécifique des prestations qui font l'objet de ces contrats nécessite, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat à long terme. Cet amendement tend ainsi à permettre aux acheteurs publics de soutenir efficacement le développement des énergies renouvelables par la promotion de nouvelles capacités de production dans les territoires, sans nécessiter de soutien de la part de l'État.

Cet amendement vise à conditionner l'entrée en vigueur de mesures contenues dans l'article 17 du présent projet de loi à la confirmation par la Commission européenne, après notification préalable, de sa compatibilité avec la réglementation L'article 17 institue des mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d'électricité. Il a notamment pour objet de permettre l'application de ce régime particulier de déduction aux charges financières nettes engagées par les sociétés de capitaux agréées mentionnées à l'article

établit des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale ayant une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. L'article en discussion instaure un plafonnement de la déduction des charges financières nettes des entreprises au montant le plus élevé entre 30 % de leur résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements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

du même code. Ce dispositif permet aux entreprises concernées de pratiquer dès l'année de réalisation de l'investissement un amortissement fiscal exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital de ces sociétés. Il s'applique dans les limites prévues par les règles européennes en matière d'aides d'État, dites règles. L'article 17 du présent projet de loi vise à réactiver ce dispositif incitatif, qui constitue l'une des mesures prévues en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d'électricité.

ni dans l'article 17 du projet de loi. Je ne suis pas favorable à un tel bornage jusqu'à 2028, pour deux raisons. Premièrement, les sociétés de financement de long terme ont besoin de temps, et une application de la déduction pendant cinq ans pourrait être

Compte tenu de leur taille, les sociétés exploitant un site éolien répondent généralement à la définition des petites entreprises au sens du code de commerce. Et dans les conditions autorisées, ces entreprises font systématiquement appel à l'option de confidentialité en application du même code, de sorte qu'à ce jour, une grande majorité des sites, notamment tous ceux qui ne sont pas détenus par des filiales de groupes français, font appel à cette option de confidentialité. Les pouvoirs publics se sont émus du résultat net consolidé dégagé par le groupe TotalEnergies, alors que ce résultat net n'a atteint que 7,6 % rapporté au chiffre d'affaires. Or les profits dégagés par les producteurs d'électricité d'origine renouvelable peuvent représenter des taux de rentabilité quatre à cinq fois supérieurs. Compte tenu de l'organisation du marché, avec l'entrée en vigueur des PPA, un producteur d'électricité renouvelable n'est pas soumis à une concurrence classique du fait du privilège d'accès au réseau dont il bénéficie.

Certaines régions de France concentrent une part importante des parcs éoliens- nous l'avons bien vu au cours de nos débats -ou photovoltaïques, du fait de conditions naturelles plus propices. Les dispositifs actuels de soutien de l'État ne permettent pas de prendre en compte les disparités régionales, comme le gisement éolien ou solaire. Cela conduit à des différences de rentabilité notable entre le nord et le sud de la France. Il est pourtant nécessaire que les projets de production d'énergies renouvelables soient répartis de façon la plus équilibrée possible, à la fois pour que chaque territoire puisse contribuer directement à une transition énergétique locale, mobilisatrice et durable, et pour éviter l'effet de saturation des riverains par la concentration de projets de grande ampleur. C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'une modulation tarifaire, en précisant que les décrets fixant les modalités d'application du tarif de rachat et du complément de rémunération seront ajustés afin de viser une répartition équilibrée des installations de production d'énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire. Quel

l'amendement n° 239 rectifié. Cet amendement vise à rationaliser le cadre d'intervention des collectivités en matière de production d'énergies renouvelables. Il a donc pour objet de rappeler expressément dans la loi que les collectivités sont pleinement habilitées à intervenir en matière d'énergies renouvelables dans le cadre des différents dispositifs prévus pour faciliter leur développement et leur financement, leurs interventions dans ce domaine ne devant en aucun cas être assimilées à une mission de service public à

à des communautés d'énergie renouvelable ou à des sociétés de production d'énergie renouvelable. De plus, nous avons prévu à l'article 18 du projet de loi que les maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale se voient proposer une participation par les sociétés de financement des énergies renouvelables situées sur leur territoire.

des installations photovoltaïques, principalement sur des toitures et des ombrières, se trouvent confrontées au choix du cadre budgétaire à respecter et à la question de savoir si la production photovoltaïque constitue ou non un service public industriel et commercial. sa décision du 29 avril 2010, le Conseil d'État considère que seules présentent le caractère d'ouvrages publics, au sens où elles sont directement affectées à un service public, les installations de production d'électricité de plus de 40 mégawatts, soit une puissance très importante- près de 30 hectares de panneaux photovoltaïques ou 15 éoliennes modernes - qui n'a aucune chance, sauf exception, d'être atteinte par un projet porté par une collectivité locale. Face à cette incertitude, les collectivités qui décident d'adopter la position la plus prudente, à savoir la création d'une régie et d'un budget annexe, se heurtent à des difficultés administratives rédhibitoires, comme la nécessité de recruter une personne externe à la collectivité pour diriger pour diriger la régie, le suivi budgétaire spécifique qui nécessite de nombreuses délibérations ou la limitation du reversement des bénéfices de l'activité dans le budget général. Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire de lever la contrainte qui pèse sur les collectivités locales souhaitant participer activement à la transition énergétique en les extrayant du cadre inadapté de la régie et du budget annexe.

Il prévoit en effet, en son 1°, que les rabais sur les factures d'électricité, décidés à la convenance du Gouvernement et imposés aux fournisseurs, seraient remboursés à ces fournisseurs par l'État. Il est donc contraire à la loi organique du 1 août 2001 sur les lois de finances (Lolf), qui prévoit, en son article 1, que les lois de finances déterminent les charges de l'État. Le 2° de l'article 18 est inséparable du 1°, car on voit mal, en équité et en droit, comment l'État pourrait ordonner à des entreprises de consentir des rabais à leurs clients sans les prendre à sa charge. Le Conseil d'État a émis des réserves sur cet article, qui ne pourrait prendre place que dans une loi de finances, fixant le montant des rabais et ouvrant un crédit, reconduit explicitement ou modifié chaque année. À vrai dire, la meilleure solution du très sérieux problème des voisins des éoliennes ne consiste pas à bouleverser leur cadre de vie tout en leur offrant des compensations financières, qui seraient souvent sans commune mesure avec les nuisances subies et pourraient varier de manière imprévisible, voire disparaître d'une année à l'autre. La vraie solution consiste à relever la distance minimale, notoirement

et 446, n'est pas souhaitable. Tout d'abord, la commission a corrigé le dispositif de partage territorial de la valeur, qui consiste en un rabais tarifaire sur la facture d'électricité lié aux installations de production d'électricité renouvelable, pour en limiter les les effets de bord. Nous avons en effet préféré une redistribution publique et collective, les communes ou leurs groupements, à une redistribution privée et individuelle portant sur l'ensemble des clients. Car les communes ou leurs groupements sont les fers de lance de la transition énergétique dans nos territoires. À l'inverse, le dispositif initial aurait conduit à une concurrence, voire à des conflits, selon que les clients sont favorables ou non à l'installation et bénéficient ou non du remboursement. Plus grave encore, la facture d'électricité n'aurait plus été la même sur l'ensemble du territoire communal, au mépris du principe de péréquation tarifaire, qui garantit un même prix de l'électricité à tous les Français. De plus, nous avons préféré un champ ouvert à toutes les énergies renouvelables, y compris le gaz ou la chaleur renouvelable, plutôt qu'à certaines d'entre elles, dans un souci de neutralité technologique. Enfin, nous avons prévu que les communes ou leurs groupements rendent compte du montant et de l'utilisation du versement, dans leur documentation budgétaire et dans leur planification énergétique. Par conséquent, le dispositif est désormais bien encadré. il n'est pas inédit, puisqu'un dispositif similaire a été appliqué à l'hydraulique et au nucléaire dans les années 1980. Le supprimer en cette période de crise énergétique reviendrait à priver les communes ou leurs groupements de recettes précieuses. Plus encore, la commission a intégré deux autres mesures complémentaires à l'article 18. D'une part, elle a prévu que l'État pourra appliquer une contribution territoriale de la valeur, c'est-à-dire un engagement au financement direct ou indirect de projets locaux, comme un critère de sélection des projets d'énergies renouvelables

issu de la commission, qui a deux mérites : corriger les effets de bord du rabais tarifaire et instituer deux compléments, sur les critères de sélection des appels d'offres et sur les modalités de constitution des sociétés de financement. C'est toute la chaîne de valeur des projets d'énergies renouvelables qui serait ainsi responsabilisée les fournisseurs, s'agissant du rabais tarifaire, les producteurs, concernant les appels d'offres, et les financeurs, pour ce qui est des sociétés de financement. Un dernier mot sur l'argument relatif à la LOLF : celle-ci n'interdit pas la création de charges dans d'autres textes que le projet de loi de finances, et ce d'autant moins que les charges visées ici et introduites par le Gouvernement lui-même seraient d'un faible montant et ne s'appliqueraient pas dès cette année budgétaire. La commission demande donc le retrait des amendements n46

Vial. Cet amendement, présenté par ma collègue Christina Pluchet, vise à faire en sorte que les rabais sur les factures d'électricité décidés à la convenance du Gouvernement et imposés aux fournisseurs soient remboursés à ces fournisseurs par l'État.

La commission des affaires économiques a, sur proposition du rapporteur pour avis, étendu le dispositif de partage territorial de la valeur, prévu à l'article 18 du projet de loi, à l'ensemble des énergies renouvelables. Par cohérence, cet amendement vise à préciser que les fournisseurs de gaz naturel, et non pas uniquement les fournisseurs d'électricité déduisent le versement d'un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situées les installations de production d'énergie renouvelable.

Cet amendement vise à calculer le versement forfaitaire, prévu à l'article 18 du projet de loi, proportionnellement aux revenus générés par les installations de production d'énergie renouvelable en lieu et place d'un calcul en fonction de la puissance installée, afin d'instaurer un véritable partage de la valeur. Corbisez. Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la disposition à la préservation du foncier agricole, alors que le développement des énergies renouvelables engendre des conflits d'usage de la terre ou des modifications de la qualité des sols. L'amendement Corbisez. Cet amendement vise à instaurer une évolution annuelle du montant du versement du partage territorial de la valeur des énergies renouvelables

des affaires économiques ? La proposition aux riverains de parts gratuites du capital des sociétés de production d'énergies renouvelables n'est pas souhaitable. En premier lieu, l'amendement est largement satisfait par le texte, puisque l'article 18 prévoit que les maires des communes et présidents des groupements d'implantation se voient informer de la possibilité de prendre une part lors de la constitution ou de la cession du capital des sociétés de production d'énergies renouvelables. Dans le même esprit, l'article 18 prévoit que ces sociétés proposent de telles parts aux riverains, aux collectivités territoriales et groupements de communes ou aux entreprises concernées.

Cet amendement vise à renforcer le dispositif de prise de participation des communes ou des EPCI aux sociétés de production d'énergies renouvelables, en fixant à deux mois le délai au terme duquel le silence apporté par ces communes ou EPCI à une demande de participation vaut refus.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Madame la ministre, mes chers collègues, il est minuit passé. Je vous propose de prolonger notre séance, afin d'achever l'examen de ce texte.

un amendement rédactionnel,

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est ouvert.